La séance est reprise.

Permettre aux agriculteurs d'avoir une véritable vision à long terme de leurs revenus, c'est mieux les protéger contre la volatilité des prix et les révisions abusives. change la logique actuelle en érigeant la contractualisation écrite en principe. Toutefois, celle-ci n'est pas toujours pertinente et c'est à à juste titre que cet article intègre la possibilité de prévoir, par un décret en Conseil d'État, un seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel les producteurs et les acheteurs peuvent y déroger. Cependant, producteurs et acheteurs ne répondent pas nécessairement aux mêmes caractéristiques. C'est pourquoi nous proposons de permettre au pouvoir réglementaire de fixer plusieurs seuils ouvrant droit à une dérogation au principe de contractualisation écrite.

non seulement en cas de calamité agricole, mais aussi en cas d'aléas sanitaires exceptionnels. Il est en effet inadmissible de faire endosser à l'agriculteur des événements indépendants de sa volonté. Pour autant, je m'interroge sur la portée de ces aléas. L'objet de l'amendement adopté en commission fait référence aux crises sanitaires relatives aux animaux, telles que la grippe aviaire ou

Même si les agriculteurs ont été très réactifs durant la pandémie que nous venons de vivre, la maladie touchant les salariés agricoles ou les conditions de circulation restreinte ont pu affecter les délais de livraison ou désorganiser la production. Il ne faut négliger aucune faille. Quel est l'avis de la commission ? Autant

autant il me semble risqué de prévoir qu'aucune pénalité ne puisse être infligée en cas de pandémie. Toute pandémie n'entraîne pas forcément une désorganisation de la production et de la récolte. En revanche, lorsqu'un producteur

Toutefois, lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, les députés ont souhaité répondre au blocage de la publication d'indicateurs faisant référence au sein de plusieurs organisations interprofessionnelles. En cas d'absence de publication d'indicateurs par une organisation interprofessionnelle, la mission serait désormais confiée à un institut technique agricole.

Elle n'a pas davantage permis un rééquilibrage durable de la répartition de la valeur ajoutée par ceux qui produisent. La question de leur juste rémunération, qui reste posée, est une question de justice sociale et de dignité.

il n'existe à ce jour aucun standard normalisé du calcul de ce même coût. Aussi, pour éviter que la prise en compte des indicateurs de coût de production ne soit anecdotique,

salariée. Cette disposition s'inscrit totalement dans les objectifs de cette proposition de loi, qui vise à donner aux agriculteurs les moyens de vivre dignement de leur métier et à reconnaître leur investissement

que, « dans le contrat ou dans l'accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle

de FranceAgriMer, des instituts techniques agricoles et des interprofessions. Il s'agit d'éviter que l'acheteur, en position de force, n'impose un indicateur qui soit source de déséquilibre dans la fixation d'un prix juste payé au producteur.

peuvent être fortement déséquilibrés et affecter la construction d'indicateurs. Une interprofession n'est pas une coalition de bienfaiteurs ni une coopérative d'associés visant à lutter pour la justice dans le monde agricole, c'est aussi un ensemble de rapports de force.

Les indicateurs de coûts de production utilisés dans les contrats ont un caractère universel, objectif et indiscutable afin d'être légitimes et crédibles. C'est le fondement d'une contractualisation engagée sur des bases solides, laquelle permettra une juste répartition de la valeur entre les acteurs. Pour cela, il est essentiel que les indicateurs de coûts de production, de marché et de qualité proviennent des organisations interprofessionnelles, lieux d'échanges et de consensus entre les différents maillons des filières. C'est pourquoi la loi doit être ferme en ce sens, en indiquant que les interprofessions diffusent des indicateurs aux opérateurs. Ce sont ces indicateurs qui doivent ensuite être utilisés dans les contrats. En effet, il n'est pas cohérent que des opérateurs disposant d'indicateurs dans leurs filières en utilisent d'autres, qui n'ont pas reçu l'aval de l'ensemble de la filière. À défaut d'indicateurs élaborés par les interprofessions, les instituts techniques agricoles, qui ont toutes les bases de données nécessaires, définissent et mettent à disposition des indicateurs.

Malgré la fin des surplus communautaires et bien que nous devions désormais importer du sucre pour équilibrer le bilan communautaire, la filière ne parvient pas à faire passer les hausses de prix- et c'est le sucre d'importation qui en profite.

Actuellement, les contrats de vente de sucre ne peuvent ni être indexés ni inclure des clauses de revoyure, car la filière n'a pas d'indicateurs de référence à disposition. Si elle était en mesure de diffuser de tels indicateurs, et ainsi de les officialiser

Dès lors, il semble nécessaire, sans pour autant supprimer l'exemption betteravière, de favoriser l'émission d'indicateurs du prix du sucre par l'interprofession afin d'encourager leur utilisation par les intervenants de la seconde transformation et de la grande distribution. Quel

me semble que c'est aussi le moment de rééquilibrer les relations entre acteurs du négoce et producteurs viticoles. Malgré les engagements contractuels, comme vous le savez très bien, le vin vendu n'est retiré qu'au bon vouloir du négoce, avec paiement soixante jours après retiraison. Les viticulteurs sont contraints de supporter les frais de stockage de vin durant de longs mois. Plus surprenant encore, certains négociants attendent la vendange suivante, lorsque les caves sont pleines et les viticulteurs en situation de faiblesse, pour imposer des réductions de prix. Parfois, ils annulent même purement et simplement les commandes, faisant ainsi fi des contrats initiaux.

Cet amendement vise à rendre automatique la saisine du ministre de l'économie par le médiateur des relations commerciales agricoles pour faire constater la nullité d'un contrat jugé illicite. Cette procédure doit en effet être améliorée afin de gagner en efficacité et en temps face au caractère périssable des produits concernés par les contrats. Il nous semble donc impératif, comme l'atelier 7 des États généraux de l'alimentation l'avait proposé, de mettre

bas. L'article L. 442-7 du code de commerce dispose que, pour caractériser un prix de cession abusivement bas, il est « notamment » tenu compte des indicateurs de coûts de production. Cet amendement a pour objet de substituer au mot « notamment », sur lequel la grande distribution peut considérablement jouer, le mot « exclusivement ». En effet, l'ordonnance du 24 avril 2019, issue de l'article 17 de la loi Égalim 1, avait pour ambition d'élargir aux produits agricoles et aux denrées alimentaires l'interdiction de céder à un prix abusivement bas, tout en supprimant l'exigence liée à l'existence d'une situation de crise conjoncturelle. Elle avait aussi pour effet de préciser les modalités de prise en compte d'indicateurs de coûts de production en agriculture. Toutefois, Toutefois, ce mécanisme demeure peu utilisé, car la notion de prix abusivement bas reste trop floue. C'est pourquoi il est nécessaire de préciser ce dispositif en fondant l'appréciation du prix abusivement bas sur les indicateurs du coût de production. choix conduirait également, en pratique, à fixer une sorte de prix plancher, en dessous duquel les acheteurs ne pourraient pas acquérir de produits agricoles sous peine de voir leur responsabilité engagée. C'est précisément le sens de notre amendement.

non seulement la Confédération paysanne, mais aussi l'UFC-Que Choisir, il est impératif d'étendre la notion de prix abusivement bas aux produits importés.

une politique de concurrence qui prévaut sur toutes les autres politiques communautaires. Il serait naïf de nier que certains distributeurs passent par des plateformes implantées à l'étranger pour contourner la loi Égalim. En ce sens, les produits agricoles importés restent le point faible de cette législation.

notre groupe et d'autres groupes politiques souhaitent en savoir plus sur l'articulation entre le chèque alimentaire durable, la rémunération des agriculteurs et la relocalisation de l'alimentation, ainsi que sur le calendrier de mise en oeuvre

C'est pourquoi cet amendement vise à préciser que la borne minimale du tunnel de prix couvre les coûts de production afin de garantir un revenu minimal à l'agriculteur : on y revient. Il s'agit de renforcer l'expérimentation de ce dispositif

afin qu'ils s'en saisissent facilement pour l'établissement des clauses de prix dans tel ou tel contrat. Limiter cette publication à certains indicateurs pertinents remet donc en cause l'efficacité de ces dispositions. C'est pourquoi nous proposons de revenir à la publication de l'ensemble des indicateurs.

liée aux matières premières agricoles afin de la rendre non négociable. Pour permettre au distributeur de connaître la part du tarif liée aux matières premières agricoles, l'article 2 offrait initialement trois possibilités

agrégée des matières premières agricoles. Il s'agit là du même niveau d'informations nécessaire pour sanctuariser les matières premières agricoles en appliquant le principe de non-négociabilité. La commission a préféré supprimer l'option 1,

Le seuil de 25 % est sans doute perfectible à bien des égards, mais il ne doit pas être rayé d'un trait de plume. Sachez qu'il ne sort pas du chapeau : il a été le fruit de concertations avec les professionnels du secteur. Nous souhaitions non seulement que le plus grand nombre de matières premières soient concernées par le dispositif, mais aussi que ce dernier soit applicable et simple d'utilisation. Il s'agissait d'un choix cohérent, visant à centrer le dispositif sur les produits alimentaires

de produits. Une concertation avec les filières devait être menée afin de préciser les produits et catégories de produits concernés. La commission des affaires économiques a choisi de supprimer ce seuil, considérant qu'il n'était pas cohérent d'inclure dans ce dispositif une soupe aux trois légumes alors qu'une soupe aux neuf légumes en serait exclue. J'entends parfaitement cette remarque : le Sénat peut précisément modifier le dispositif

alors que notre volonté première est de cibler ceux qui utilisent vraiment des produits agricoles. Je ne suis pas sûre qu'il soit utile de favoriser les grandes firmes. Bref, discutons, menons des concertations. Travaillons à un dispositif qui puisse comprendre un seuil de matières premières, mais ne nous contentons pas d'une suppression sèche.

Ce que la commission propose, c'est de supprimer la liste détaillée, de conserver la liste agglomérée et d'ajouter, au même niveau, le tiers de confiance.

apporter de la transparence permet une revalorisation des prix sur les produits à forte composante agricole auprès de la grande distribution- en intégrant, bien sûr, le coût de production des matières

Cet amendement vise à encadrer les modalités d'adoption du décret. La publication de ce décret doit être précédée d'une concertation et d'un avis favorable de l'interprofession. De plus, il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations. De nombreuses filières ou de nombreux maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d'application de l'article 2. Il semble important de signifier dans le texte que l'accord de tous est requis pour qu'un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l'article. La parole est à Mme Corinne Imbert,

La construction du prix des vins et spiritueux n'est que peu liée au coût des matières premières. C'est le coût du travail, de la transformation et du développement des marques qui compte dans la valeur du produit. S'agissant tout d'abord du secteur vitivinicole, celui-ci est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. Pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an après la récolte ou au début de la campagne viticole. Les prix ne fluctuent donc pas comme dans d'autres filières et il n'est pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix en aval dans les conventions annuelles, puisque les prix des matières premières agricoles n'évoluent pas en cours d'année.

de celui-ci. Dès lors, qu'il s'agisse des vins ou des spiritueux, il paraît peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur.

d'une concertation ou d'un avis de l'interprofession pour éviter toute sortie abusive. En effet, de nombreuses filières ou de nombreux maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d'application de l'article 2. Il semble important de préciser que l'accord

des filières puisse participer à cet effort. C'est une demande de la plupart des organisations représentatives des exploitants agricoles. Comme Franck Menonville l'a rappelé, le texte prévoit cependant un champ d'exclusion pour un certain nombre de produits alimentaires dont la liste serait définie par

ou à la filière viticole, il faut prévoir pour d'autres produits que les opérateurs justifient leur demande de dérogation. L'avis de l'interprofession doit être un préalable.

cet amendement a pour objet d'inclure dans la rédaction du décret l'objectivation des difficultés rencontrées par les opérateurs et les spécificités causales validées par l'interprofession. L'accord de tous doit être requis pour qu'un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par la

est tenu par le contrat écrit qu'il devra désormais souscrire et qui le liera directement à l'agriculteur. Lorsqu'il obtiendra une revalorisation du tarif auprès du distributeur, celle-ci découlera de la

à laquelle nous nous opposons, est réintroduite.

en revanche, placer les industries agroalimentaires et les transformateurs- les petits comme les grands -en situation de fragilité par rapport à la distribution.

il est nécessaire que les évolutions des coûts et des matières premières soient prises en compte dans la construction du prix, du premier jusqu'au dernier maillon de la chaîne de valeur. Cela ne peut s'envisager sans une révision des modalités de détermination du seuil de revente à perte (SRP). (SRP). Il s'agit donc de revoir les modalités de ce seuil en excluant des autres avantages financiers consentis par le vendeur les rémunérations perçues par le distributeur au titre des services de coopération commerciale ainsi que celles qui sont obtenues en contrepartie

Cet amendement, travaillé avec des professionnels du monde agricole, vise à compléter le dispositif de renforcement du respect du tarif de l'industriel. Celui-ci ne peut discriminer un distributeur par rapport à son tarif qu'à la seule condition d'obtenir, pour chaque dérogation sous forme de réduction de prix, de prix, une contrepartie réelle et proportionnée, conformément aux dispositions du code de commerce. Une telle disposition renforcerait par ailleurs la traçabilité de la construction du prix, en partant du tarif de l'industriel pour parvenir au prix convenu. Conformément à la loi, les conditions générales de vente de l'industriel doivent être le socle de la négociation commerciale, ce qu'elles ne sont plus depuis longtemps. Elle faciliterait ainsi également les contrôles du respect du formalisme par l'administration. En cela, elle participerait à l'objectif de transparence. Il s'agit d'incorporer dans le code de commerce la proposition n° 33 du rapport de la commission d'enquête parlementaire sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs, qui s'est achevée le 25 septembre 2019. Cette proposition vise à répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs et à établir un barème des prix exigés pour ces services. Les fournisseurs sont astreints à une obligation légale de transparence sur les prix proposés dans leurs conditions générales de vente. La réciprocité imposée aux distributeurs en matière de services proposés aux fournisseurs ne peut être que vertueuse, en donnant toute transparence sur les prix pratiqués en la matière, en évitant toute discrimination injustifiée et en permettant d'apprécier la proportionnalité entre ces services et les sommes exigées en contrepartie.

le calcul du SRP. Cela aurait pour conséquence d'augmenter fortement les prix à la consommation de tous les produits, pas seulement des produits alimentaires, puisque, désormais, le distributeur devrait proposer un prix de vente comme s'il n'avait proposé aucun service commercial en contrepartie.

pour deux raisons. D'une part, la clause de renégociation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est-à-dire fondée sur l'évolution du prix des matières premières agricoles et de l'énergie, deviendra caduque, puisque les articles 1 et 2 de cette proposition de loi créent une clause de révision automatique des prix selon l'évolution des matières premières agricoles. Il n'y aura donc plus besoin de renégocier, la modification sera automatique.

qui serait source d'inflation et, surtout, qui serait difficile à mettre en oeuvre en raison de l'absence d'indicateurs partagés sur ces intrants comme les emballages, le transport, etc., la commission propose donc une clause de renégociation obligeant les parties à se réunir

une grande compagnie qui produit une boisson sucrée de couleur brunâtre et avec une étiquette rouge- si vous voyez ce que je veux dire ! -, ces

consiste à assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits de marque de distributeur (MDD) au même formalisme contractuel que les produits de marque. Il s'agit de préciser les mentions de la convention unique prévues dans le code de commerce à propos des engagements convenus entre la grande distribution et ses fournisseurs pour la fourniture de produits sous marque de distributeur en prévoyant l'insertion systématique de clauses relatives au chiffre d'affaires prévisionnel, aux volumes, à l'innovation. Conformément à l'obligation consacrée dans le code de commerce, il convient également de rendre obligatoires la réponse du distributeur à la suite de la réception des conditions générales de vente ainsi que la mention des conditions générales de vente dans le contrat de fourniture.

Nous avons en effet intégré, dans les contrats de MDD, une durée minimale, une clause de révision automatique des prix, une obligation d'informer le fabricant en amont si le volume prévisionnel risque de ne pas être respecté, une durée minimale de préavis, une clause de répartition des coûts ainsi que l'interdiction de mettre à la charge du fabricant les dépenses de promotion. Il s'agit d'un encadrement inédit, qui permettra d'inclure l'ensemble du secteur alimentaire dans la poursuite de l'objectif d'une meilleure rémunération des agriculteurs

parole est à Mme Patricia Schillinger. Alors que les produits de marques de distributeurs occupent une place croissante dans les rayons et constituent un réel débouché pour les productions

Tout d'abord, il vise à ce que l'appel d'offres ou le contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires comporte impérativement un engagement sur des volumes prévisionnels. Les agriculteurs pourront ainsi disposer d'une vision de long terme sur leurs revenus à venir. Cet amendement tend également à introduire une clause de révision automatique des prix résultant du coût de la matière première agricole dans les contrats portant sur la conception et la production de produits alimentaires.

Cet article vise à une meilleure information du consommateur sur la juste rémunération du producteur. À ce titre, la cascade des indicateurs du contrat amont vers le contrat aval n'est aujourd'hui pas suffisamment appliquée. L'acheteur de produits agricoles est pourtant soumis à cette obligation, prévue dans le code rural et dans le code de commerce. Au regard de la complexité de certaines chaînes d'approvisionnement dans les différentes filières agricoles, il convient donc de renforcer cette cascade. Cet amendement a ainsi pour objet de prévoir que les indicateurs soient contenus dans la clause de prix du contrat passé entre l'acheteur de produits agricoles et son propre client.

soumis à l'interdiction du seuil de revente à perte ni aux dispositions de l'article 2, puisque les fournisseurs proposent rarement des conditions générales de vente à leur distributeur. L'esprit du système de la cascade doit donc être renforcé par rapport à la rédaction issue de la loi Égalim pour les produits MDD. La parole

vise à proposer un cadre pour l'intervention du tiers indépendant en ce qui concerne la clause de révision automatique des prix. Désormais, le tiers devra attester de la véracité des informations sous quinze jours.

La commission des affaires économiques a effectué un pas dans la bonne direction en renforçant l'article 2 B. Cependant, prévoir pour le distributeur une obligation d'engagement sur un volume prévisionnel dans le cadre d'un contrat MDD ne semble pas suffisant. C'est en effet sur des volumes réels, et pas seulement sur des volumes prévisionnels, que le contrat devrait comporter un engagement. le fournisseur de produits à marque de distributeur engage des investissements non seulement pour produire des MDD, mais aussi pour les concevoir. Il semble donc plus difficile pour le fabricant de MDD de fixer un prix juste, rémunérateur pour les producteurs s'il n'a pas de visibilité sur les volumes. Le présent amendement vise donc à imposer au distributeur un engagement sur les volumes lors de la signature d'un contrat conclu avec son fournisseur. Celui-ci portera sur la conception et la production de produits vendus sous marque de distributeur.

n° 121 rectifié est partiellement satisfait. En commission, nous avons veillé à prévoir que l'acheteur doit prévenir le plus tôt possible le fabricant s'il a connaissance que des faits l'empêcheront de respecter les volumes prévisionnels. En revanche, nous considérons qu'il n'est pas obligatoirement que tous les coûts additionnels seront à la charge du distributeur, car cela dépend bien entendu de la nature de ces coûts additionnels. L'important reste surtout que le fabricant n'ait pas de surprise en cours d'exécution.

En effet, dans le même esprit qu'à l'article 2, il convient de préciser ce que nous entendons par « tiers de confiance » ou « tiers indépendant », afin qu'il n'y ait pas de contentieux sur le sujet. Quel est l'avis du Gouvernement

modifié. bis B Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est minuit ; je vous propose de prolonger la séance jusqu'à minuit et demi afin de poursuivre plus avant l'examen de ce texte.

dans les contrats, afin de prévoir une marge d'erreur suffisante et conforme à la réalité de la vie économique actuelle. Les taux de service actuellement imposés par les distributeurs sont en moyenne autour de 98,5 % et peuvent atteindre 99,9 % dans des cas extrêmes. Ces situations fortement regrettables génèrent l'application de pénalités qui deviennent quasiment automatiques. Si la rédaction actuelle de l'article 2 C offre un début de réponse en prévoyant « une marge d'erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévu par le contrat elle renvoie néanmoins à un décret le soin de fixer le taux. Le présent amendement vise à s'assurer que ce futur décret s'inscrive bien dans l'esprit de la loi, à savoir la fixation d'un taux réaliste et adapté à la vie économique.

Il s'agit de s'assurer d'une application juste et proportionnée des sanctions et d'éviter ainsi les nombreux abus auxquels nous assistons actuellement et dont les fournisseurs sont les uniques victimes. En effet, la réciprocité avec la grande distribution n'a aucune existence aujourd'hui. Plus concrètement, nous estimons que si aucune perte de chiffre d'affaires n'est enregistrée, rien ne justifie d'appliquer des pénalités aux fournisseurs. Il est trop fréquent que les pénalités logistiques deviennent des sources de profit à part entière pour la distribution, ce que nous combattons farouchement. L'amendement n° 32, présenté Tissot. Cet amendement tend également à préciser la rédaction de l'article 2 C. Il vise à prévoir explicitement que lorsqu'un état d'urgence sanitaire est déclaré, aucune pénalité logistique ne peut être infligée. Il apparaît en effet que malgré le caractère exceptionnel de la situation liée à la crise de covid-19, certaines enseignes, insatisfaites d'un taux de service inférieur aux standards habituels dont elles sont pourtant par ailleurs partiellement responsables, ont remis en vigueur des pénalités logistiques sans commune mesure avec le préjudice économique subi. si la rédaction de l'article 2 C prévoit que, en cas de force majeure, de telles pénalités ne pourront pas être infligées, et malgré le fait que Mme la rapporteure nous a indiqué en commission que notre amendement était satisfait, nous estimons indispensable de préciser que la déclaration d'un état d'urgence sanitaire constitue automatiquement

Si un contrat est mal exécuté par un industriel, il se peut que le distributeur subisse tout de même un préjudice, qui peut être de notoriété, par exemple, si les rayons sont remplis, mais que le produit ne se révèle pas conforme aux exigences sanitaires.

Il est inscrit noir sur blanc à l'article 2 C que les pénalités sont interdites en cas de force majeure et qu'il doit toujours être tenu compte des circonstances indépendantes des parties.

selon son contenu et la date de son application, sous réserve d'une information du client dans un préavis d'au moins trois mois. Cette mesure n'atteint aucunement le principe de négociabilité des conditions commerciales entre fournisseur et distributeur ni la liberté du distributeur de référencer ou non telle gamme de tel fournisseur en fonction de la demande et des offres concurrentes. À l'instar de l'agriculteur qui sera en capacité d'imposer des hausses de prix, à l'instar du distributeur qui a la pleine maîtrise de ses prix au consommateur, le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l'année, sans risque que la loi ou le contrat ne fige un « prix convenu » pour le temps de la convention récapitulative. Cette mesure est le complément nécessaire de l'impérative application de l'évolution des prix des matières premières agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d'une réelle répartition de la valeur au sein de la filière de l'amont vers l'aval. Seul le respect des prix agricoles et des tarifs du transformateur permettra d'inverser durablement le mécanisme de formation des prix en partant de l'amont. Enfin, eu égard à l'interdépendance de la filière, cette mesure est l'élément indispensable pour renforcer les transformateurs PME qui privilégient l'approvisionnement local et les circuits courts. Elle contribuera ainsi à rééquilibrer leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution. Vous l'aurez compris, cet amendement a pour objet de soutenir les PME agroalimentaires françaises, ancrées dans les territoires, qui pourraient se trouver de fait exclues des négociations des contreparties pertinentes.

proposition de loi est, selon le rapporteur, une « fusée à plusieurs étages ». Au-delà du travail de construction du prix en amont en faveur des agriculteurs, la relation industriel-fournisseur mérite aussi toute notre attention. N'oublions pas que notre territoire est irrigué par de nombreuses PME agroalimentaires qui doivent faire face à la pression des distributeurs pour des prix à la baisse. Le transformateur doit donc pouvoir conserver une certaine maîtrise de son tarif. C'est ce à quoi tente de répondre l'article 2D, que nous proposons de compléter.

Cet amendement vise donc à rééquilibrer les relations entre les fournisseurs et les distributeurs en introduisant un mécanisme qui garantisse qui garantisse l'adaptabilité réelle et continue des prix pratiqués par les fournisseurs à leurs clients-distributeurs, tout au long de l'année, afin de prendre en compte les variations des coûts agricoles et de transformation. Il s'agit de rendre impérative l'application homogène du tarif général du fournisseur selon son contenu et la date de son application, sous réserve d'une information du client dans un préavis d'au moins trois mois. Avec ces nouvelles mesures, l'agriculteur sera en mesure d'imposer des hausses de prix, tandis que le distributeur conservera la pleine maîtrise de ses prix au consommateur. Le transformateur doit pouvoir maîtriser son tarif général tout au long de l'année, sans risque que la loi ou le contrat ne fixe le prix convenu pour le temps de la convention récapitulative. Cette mesure est le complément nécessaire de la non-négociabilité des prix agricoles. Elle crée et assure ainsi les conditions d'une réelle répartition de la valeur au sein de la filière, de l'amont vers l'aval. Enfin, cette mesure permettrait de renforcer les transformateurs PME, qui font souvent plus d'effort que les grands groupes pour privilégier l'approvisionnement local et les circuits courts dans leur rapport de force très déséquilibré avec la grande distribution. Si on ne rééquilibre pas les relations entre transformateurs et grande distribution, on reste dans un rapport de force favorable pour le distributeur, qui peut pénaliser l'intégralité de la chaîne. Ces trois amendements identiques tendent à interdire absolument toute négociation sur le tarif du fournisseur, au-delà même des matières premières agricoles.

et c'est pourquoi nous avons adopté il y a quelques instants les amendements n 107 rectifié et 114 rectifié, ainsi que l'amendement n° 159 de la commission, qui permettent aux industriels de rouvrir la négociation en cas d'évolution des coûts comme l'emballage, le transport et l'énergie.

Nous avons réglé le problème de la pénalité logistique, nous avons réglé le problème du retrait-rappel, circonstance dans laquelle le distributeur demande des sommes qui sont totalement disproportionnées à la réalité des faits,

revanche, manque encore un élément : l'harmonisation de la facturation. Il n'est pas normal, aujourd'hui, que les fournisseurs soient la banque des distributeurs.

Ce que je comprends de l'amendement, c'est que si le distributeur veut se faire de la trésorerie sur le dos de son fournisseur, il fait en sorte que le délai de paiement qu'il impose à son fournisseur soit supérieur aux délais de paiement auxquels le fournisseur est lui-même soumis en amont.

apporter quelques précisions. Cela ne concerne absolument pas l'amont, mais uniquement les relations entre industriels et distributeurs. Il s'agit de faire en sorte que le distributeur ne demande pas au fournisseur de payer plus rapidement les pénalités logistiques qu'il n'a lui-même payé la livraison de la marchandise.

Gremillet, Michel Raison et de Mme Anne-Catherine Loisier rédigé au nom de la commission des affaires économiques du Sénat constatait que le relèvement du seuil de revente à perte, introduit dans la loi Égalim, a malheureusement produit des effets « pervers » pour certaines filières agricoles, notamment les producteurs de fruits et légumes Le rapport prend l'exemple de la fraise gariguette, pour laquelle, malgré la revalorisation du seuil de revente à perte de 10 %, le distributeur a souhaité maintenir son prix de vente consommateur intégrant la revalorisation obligatoire de 10 %, conformément à la loi, tout en durcissant les négociations avec son fournisseur. Dès lors, à perte (SRP) de 10 % s'est traduite, en l'espèce, par une baisse de 10 % du prix d'achat aux producteurs. La loi Égalim vient alors, à rebours de son ambition initiale, d'une part, complexifier les relations commerciales et, d'autre part, provoquer un effet déflationniste. Le présent amendement vise ainsi à mettre un terme à cet effet pervers qui pénalise les producteurs. La parole est à M. Laurent

la revalorisation de 10 % du seuil de revente à perte s'est traduite, pour les agriculteurs producteurs de fraises, de tomates, de concombres et autres, par une baisse directe d'un même montant de leur rémunération.